La séance est ouverte. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

je soumets aujourd’hui à votre examen une proposition de loi simple, univoque et laconique. Simple, car elle s’appuie sur le bon sens. Univoque, car elle clarifie la loi. Laconique, enfin, car elle tient en une seule phrase.

J’en ai beaucoup parlé avec M. le rapporteur, que je remercie de sa disponibilité. Ce texte vise à encadrer juridiquement le mariage des personnes séjournant irrégulièrement en France. Pour le dire plus simplement, il tend à ce que le mariage ne soit autorisé qu’aux personnes séjournant de manière régulière sur notre territoire.

comment se fait il que cette mesure ne soit pas déjà en vigueur ? Eh oui ! Comment est il possible de marier quelqu’un qui n’est pas en situation régulière sur le territoire ? Est il concevable de lire des articles du code civil, au sein de la maison municipale de la République, à une personne qui n’a pas le droit d’être là ? sont les retours et les réactions interrogatives de ceux à qui j’en parle. Pourtant, si cette mesure semble évidente à beaucoup, notre droit, en l’état, ne permet pas de s’opposer au mariage d’une personne en situation irrégulière

Je voudrais d’ailleurs vous rappeler l’expérience douloureuse de Stéphane Wilmotte, maire d’Hautmont, que nous avons reçu la semaine dernière au Sénat. Il avait refusé de célébrer le mariage d’un individu placé sous obligation de quitter le territoire français, ancien président d’une mosquée fermée pour discours haineux et apologie du djihad armé. ! À ce titre, notre collègue Wilmotte a reçu des menaces de mort et subi des pressions. Son domicile a dû être protégé. C’est le monde à l’envers : l’individu sous OQTF a porté plainte contre le maire, qui a de ce fait encouru une peine de prison et d’inéligibilité, ainsi que le versement de dommages et intérêts Heureusement, la justice a tranché en sa faveur. Mais comment est il possible de placer un élu de la République dans une telle situation ? Comment est il possible que les maires risquent de longs mois de procès, parfois aggravés d’un stress personnel et familial, alors qu’ils agissent pour le bien du territoire ? S’il est bien un espace parlementaire pour répondre à ces interrogations, c’est celui du Sénat. La législation actuelle contre les mariages de complaisance est insuffisante et place les officiers d’état civil dans des situations ubuesques. face à une demande de mariage émanant d’une personne en situation irrégulière, le maire doit rechercher « une présomption de fraude », ou examiner « la sincérité de l’union Bref, on lui demande de se transformer en inspecteur Colombo ou en ersatz d’huissier conjugal pour enquêter. Bravo ! Mes chers collègues, comme vous le savez, ce n’est pas le rôle du maire, d’autant plus que sa volonté d’investiguer, ou celle de l’adjoint délégué, variera selon sa propre sensibilité.

Pour le dire autrement, il n’y a pas d’égalité de traitement. Ces disparités peuvent même être interprétées comme une inégalité devant la loi, en complète opposition à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui dispose

Je souhaite également anticiper les préoccupations légitimes que soulève ce texte, notamment au regard de la protection des droits et du respect des libertés individuelles.

Pour rendre sa décision, le Conseil constitutionnel s’était fondé sur les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui consacrent la liberté personnelle. Je tiens donc à rappeler spécifiquement les termes La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme a d’ailleurs régulièrement clarifié sa position, indiquant que, concernant les restrictions que la loi nationale peut appliquer au droit du mariage, les États jouissent d’une « ample marge d’appréciation », notamment lorsqu’ils sont appelés à protéger les intérêts de la société. On pourrait d’ailleurs citer ici l’exemple du Danemark, pays membre de l’Union européenne, qui impose depuis 2002 la détention d’un titre de séjour valide pour les étrangers qui souhaitent se marier dans le pays. Même si certains devaient me rappeller la particularité danoise liée au mécanisme d’exemption, il n’en reste pas moins vrai que je ne fais que proposer la même mesure. C’est également le cas, depuis 2011, pour la Suisse, pays membre du Conseil de l’Europe. Il a raison ! Oui, mes chers collègues : le mariage est une institution protégée par la loi, mais rien n’interdit de la préciser, donc de la faire évoluer, pour éviter des contournements de son esprit. Je souhaite appeler aujourd’hui à un débat riche et constructif, ainsi qu’à l’examen approfondi des amendements déposés sur ce texte.

Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. » Mes chers collègues, il me semble que cette proposition de loi est utile et qu’elle renforce les lois de notre République.

éclairer nos collègues membres d’une autre commission en dressant un rapide état du droit en la matière. Actuellement, la liberté du mariage est, certes, consacrée

que par la loi, donc par le législateur, comme l’a rappelé, à plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel. Nous sommes donc, aujourd’hui, dans notre rôle. Les restrictions à la liberté du mariage prévues par la législation française sont cependant peu nombreuses : elles sont quatre et concernent exclusivement les mineurs, la polygamie, la consanguinité

sérieux laissant présumer » un mariage simulé ou arrangé. Le procureur a ensuite le choix de laisser

Bien que ces dispositions constituent une entrave à la liberté du mariage, le Conseil constitutionnel a considéré que le cadre législatif actuel était conforme à la Constitution. D’une part, en effet, cette liberté « ne fait pas obstacle à ce que le législateur prenne des mesures de prévention ou de lutte contre les mariages contractés à des fins étrangères à l’union matrimoniale ». D’autre part, il a réfuté explicitement l’existence d’un droit de contracter le mariage à des fins étrangères à l’union matrimoniale. Il y a donc une reconnaissance constitutionnelle de ces bornes à la liberté du mariage. Cependant, celle ci est, en l’état du droit et de la jurisprudence actuels, dissociée du droit au séjour. Autrement dit, liberté du mariage n’est pas conditionnée à la régularité du séjour. C’est la raison pour laquelle le maire, en tant qu’officier d’état civil, ne dispose d’aucun pouvoir pour s’opposer formellement au mariage de toute personne présente en situation irrégulière sur le territoire national, ou encore d’une personne soumise

du mariage […] s’oppose à ce que le caractère irrégulier du séjour d’un étranger fasse obstacle, par lui même, au mariage de l’intéressé ». Ainsi, l’officier d’état civil ne peut, en l’état actuel du droit, demander une pièce justifiant de la régularité du séjour des futurs époux, même à titre informatif. Le code pénal prévoit d’ailleurs qu’un maire qui s’opposerait, de façon illégale, à la célébration d’un mariage est passible d’une peine de

examen, la semaine dernière – pour des raisons sans doute différentes d’un groupe politique à l’autre… Il ne s’agissait toutefois pas d’un rejet sec, et cela pour deux raisons.

de toutes les informations nécessaires à l’appréciation de la légalité des mariages et, d’autre part, le renforcement de la prévention et de la lutte contre les mariages simulés ou arrangés, qui

nous avons déposé, en vue de la séance publique, des amendements de nature, selon moi, à concilier les exigences du Conseil constitutionnel et les objectifs de cette proposition de loi.

insiste, ont un caractère détachable du dispositif initial du texte. Ils peuvent être vus, soit comme tendant à le compléter utilement en précisant les moyens dont disposeront les maires et le ministère public

certains textes que nous sommes amenés à examiner exigent des démonstrations juridiques très fines. D’autres relèvent de la simple évidence, pour ne pas dire du bon sens.

la proposition de loi qui nous est présentée est nécessaire, parce qu’elle répond à une incohérence criante : comment un État peut il constater qu’une personne est en situation irrégulière, en lui permettant d’accéder à une institution aussi forte et symbolique que le mariage, qui ouvre, en droit français, des droits durables ? La situation irrégulière signifie, par essence, que l’intéressé n’a pas vocation à demeurer de manière prolongée sur le territoire national. Dans ces conditions, comment justifier l’accès à une institution qui consacre une forme de pérennité ? Par l’amour ! Cette contradiction fragilise l’autorité de l’État et nourrit l’incompréhension criante de nos concitoyens. Plus encore, elle vient placer, au cœur de ce paradoxe, les acteurs essentiels de la démocratie que sont les maires, représentants de l’État, représentants du préfet, représentants du procureur de la République.

Un mariage oblige à une communauté de vie. Un mariage oblige au secours, à l’assistance, à l’éducation des enfants

comment contribuer à une communauté de vie, au secours, à l’assistance, à l’éducation des enfants et à la pérennité de la famille quand on doit être expulsé du territoire national ? « Mariage d’amour, mariage d’argent, j’ai vu se marier toutes sortes de gens », disait Brassens. Mais les maires sont souvent les spectateurs des tentatives d’instrumentalisation de cette institution. Nous ne comptons plus les témoignages d’élus qui font part de leur malaise face à des situations où la fraude est soit criante, soit larvée, ce qui les place dans une position dans laquelle le courage n’est, aujourd’hui, plus suffisant. En l’état de notre droit, et alors même qu’ils ont connaissance de la situation irrégulière du futur conjoint, des maires se retrouvent contraints de célébrer un mariage ouvrant le droit direct à une régularisation. Quand bien même un signalement au parquet aurait été réalisé, quand bien même le parquet aurait répondu, quand bien même une mesure d’éloignement aurait été ordonnée, le maire se retrouve obligé de célébrer une union qui ne constituera qu’un obstacle à l’État de droit. Si cette proposition de loi est l’œuvre d’un sénateur, il ne faut pas y voir un hasard. Le Gouvernement et la société ne peuvent être sourds à la volonté de la chambre représentant les collectivités locales, porte parole des maires.

Mettre en cohérence notre droit est, avant tout, une manière de protéger les maires, de leur redonner les moyens d’agir face aux abus, mais, surtout, de restaurer l’autorité de l’État et la force de nos lois dans chacune des mairies de France. Remettre du bon sens dans notre droit et du bon sens au ministère de la justice, voilà le sens de l’œuvre du sénateur Demilly, que je soutiens particulièrement. Deux débats vont donc se tenir ce matin, dont la légitimité est bien sûr entière. Sur le fond, certains soutiendront que cette mesure constitue une atteinte aux libertés fondamentales. À ceux là, je veux dire très clairement que, en République, les droits s’acquièrent dans le respect des règles communes, et d’aucune autre La régularité du séjour est la condition même de l’intégration. Ainsi, permettre à une personne en situation irrégulière de se marier ouvre le droit à une régularisation, ce qui affaiblit considérablement nos règles de vie en commun, ainsi que la loi votée par le Parlement et validée par ailleurs par le Conseil constitutionnel.

Demander au Conseil constitutionnel de réexaminer sa position n’est pas un acte de défiance, mais, bien au contraire, un acte de confiance en sa capacité à s’adapter aux réalités de notre temps, comme l’ont voulu Michel Debré et le général de Gaulle en rédigeant la Constitution de 1958.

effet l’obligation, sous peine de sanction pénale, de marier une personne dont ils savent qu’elle ne respecte pas les règles du droit au séjour et pour laquelle l’autorité administrative a parfois délivré une obligation de quitter le territoire français. Le maire est alors censé se mettre des œillères et célébrer le mariage comme si de rien n’était… Non, cette règle n’est plus acceptable.

y compris si le maire a face à lui un salafiste en situation irrégulière qui prêche la haine de notre pays. Bravo ! Très bien ! Lorsque l’on décrit cette réalité juridique, nos concitoyens sont comme nous, ils sont choqués,

civil, mais d’une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a placé la liberté du mariage au dessus des règles régissant le droit au séjour en France. Il s’agit d’une interprétation du Conseil

nom de « la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789 », toutes les dispositions législatives qui feraient « du caractère irrégulier du séjour d’un étranger un obstacle, par lui même, au mariage de l’intéressé Voilà où nous en sommes en 2025, mes chers collègues : un maire ne peut pas refuser de marier une personne qui, en application de la loi française, ne devrait plus être sur le territoire national

se retrouvent aujourd’hui devant les tribunaux. Cette réalité brutale est difficilement compréhensible. Je reconnais humblement que je ne me sens capable de justifier une telle situation sur le terrain ni auprès des maires de mon territoire ni auprès de nos concitoyens.

J’espère aussi que le Sénat, en tant que chambre des territoires, soucieuse des préoccupations des élus municipaux, adoptera la proposition de loi que nous vous soumettons, J’espère enfin qu’il ne s’agira pas d’un coup d’épée dans l’eau et que le Gouvernement se saisira du texte pour le porter à l’Assemblée nationale, comme il a su le faire récemment pour d’autres propositions de loi sénatoriales, au premier rang desquelles la proposition de loi Sans surprise, les sénateurs du groupe Union Centriste voteront évidemment en faveur de ce texte. La parole

ce texte n’est pas. Ce texte ne vise pas à lutter contre les mariages blancs, gris ou arrangés, tout d’abord parce que, à l’évidence, le séjour irrégulier n’a strictement aucun rapport avec l’intention matrimoniale ou le consentement. Sauf Sauf à considérer que la situation légale d’une personne au regard de son séjour en France aurait un lien mécanique avec sa sincérité ou son honnêteté, on voit mal, même y mettant beaucoup de xénophobie, comment arriver à un tel résultat.

Il s’agit non pas de protéger le principe du mariage d’amour, mais d’empêcher les mariages d’amour lorsque cet amour implique une personne de nationalité étrangère en situation irrégulière, parce que le fait que cette personne puisse obtenir des droits en se mariant vous est insupportable

! Aujourd’hui, vous entendez priver de ces droits de nombreux couples binationaux, qui, pour beaucoup, ne pourraient plus se marier du tout, parce que l’un des époux vient d’un pays en guerre, d’un pays où le mariage est soumis à des restrictions religieuses, d’un pays où l’homosexualité est criminalisée. Pis encore, ce texte vise en réalité à aller beaucoup plus loin. Mardi dernier, et ce n’est pas un hasard du calendrier, a eu lieu l’audience de Robert Ménard, mis en examen pour avoir refusé de célébrer le mariage d’Éva et de Mustapha, un couple franco algérien, au motif que Mustapha était soumis à une OQTF. Et Robert Ménard d’expliquer au couple : « Je sais bien que ce n’est pas un mariage blanc, mais pour moi c’est un moyen de mettre le sujet des OQTF sur la table. »

qui met en péril nos politiques migratoires, ainsi que la sécurité de nos élus ». Mais quel serait donc ce fléau ? Tenez vous bien mes chers collègues, il s’agit du mariage, de l’amour entre deux êtres qui aspirent à passer le reste de leur vie ensemble

incitant les maires et les officiers d’état civil à sortir de leur seule mission, la célébration des mariages, pour devenir des acteurs du contrôle de l’immigration. Tel n’est pas leur rôle ! Leur rôle est de vérifier que le mariage est fondé sur le consentement libre et éclairé des futurs époux,

peu ! Dans sa décision du 20 novembre 2003, le Conseil constitutionnel, considérant que la liberté du mariage est une composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4

Votre amendement est contraire non seulement à nos engagements internationaux, mais également à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui s’appuie sur deux articles de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Convenez qu’il est possible de modifier beaucoup de choses, mais qu’il serait très osé – mais après tout, pourquoi pas ? – de vouloir modifier la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

il y a des femmes et des hommes. Il y a un étudiant qui est dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour. Il y a un travailleur qui vit depuis vingt ans en France et qui attend le renouvellement de sa carte de résident. Il y a Liri, cette jeune kosovare qui habite à Rouen, qui parle cinq langues

De plus, comme vous le savez, le manque cruel de moyens dans nos préfectures crée des situations ubuesques, des personnes se retrouvant dans l’irrégularité simplement parce que leur dossier n’a pas été traité en temps et en heure. Enfin, cette proposition visant à alimenter de fausses polémiques, moi de rappeler quelques faits. Le mariage ne conduit pas automatiquement et encore moins immédiatement à la régularisation. Mais ça aide ! Les démarches nécessaires sont longues et ne présentent aucune garantie d’aboutissement. Le mariage ne protège en rien d’une obligation de quitter le territoire ni d’un arrêté d’expulsion.

Ce texte est symptomatique de la dérive d’une droite qui n’a plus de républicain que le nom et qui se laisse dicter ses propositions de loi par l’extrême droite. Cette proposition de loi arrive après la mise à l’agenda de l’expression, empruntée à Jean Marie Le Pen lui même, de « submersion migratoire », après la circulaire Retailleau visant à durcir la régularisation des

pas à pas, vous démantelez nos principes fondamentaux et notre démocratie. Face à vous, nous demeurons les seuls garants des valeurs républicaines. Non, vous les détruisez ! Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste votera contre ce texte, qui est contre la Constitution et contre l’amour.

à une faille législative qui fragilise notre souveraineté, affaiblit notre État de droit et met en danger nos élus locaux. Chaque année, près de 230 000 mariages sont célébrés dans notre pays. Un certain nombre d’entre eux implique un conjoint en situation irrégulière sur le sol français. Ce phénomène est une brèche béante dans notre législation, qui permet à des étrangers illégaux de contourner les règles de notre politique migratoire. Comment justifier qu’un individu qui ne respecte pas nos lois en matière de séjour puisse revendiquer un droit aussi fondamental que le mariage républicain,

Aujourd’hui, ils sont contraints de célébrer les mariages, y compris lorsqu’ils savent que l’un des époux réside illégalement dans notre pays. Le maire d’Hautmont a par exemple demandé le report de la célébration du mariage d’un homme sous obligation de quitter le territoire français qui était l’ancien président d’une mosquée fermée pour radicalisation par le ministre de l’intérieur. Que s’est il passé ensuite ?

Autre exemple marquant, Robert Ménard, maire de Béziers, a également pris position contre ces mariages de complaisance, qui sont devenus une véritable industrie. Il a dénoncé publiquement des cas où des personnes en situation irrégulière tentaient de régulariser leur statut le mariage, souvent avec des complicités. Faut il rappeler qu’un tiers des OQTF ne sont jamais exécutées ? En facilitant ces unions, nous entretenons un système dévoyé et inefficace, mes chers collègues. Il nous faut au contraire donner à nos maires et à nos élus locaux les outils nécessaires pour défendre la République et cesser de les exposer à des représailles lorsqu’ils agissent avec courage et bon sens. Le Rassemblement national soutient avec force cette proposition de loi, qui s’inscrit pleinement dans notre combat contre l’immigration incontrôlée et l’impunité dont bénéficient ceux qui violent nos lois. Depuis des années, nous dénonçons ces détournements du droit qui affaiblissent notre souveraineté et font peser une charge supplémentaire sur notre nation.

Loin d’une atteinte aux droits fondamentaux, c’est une mesure de bon sens, d’ordre et de justice. Nous avons le devoir d’agir pour mettre fin à ce laxisme qui mine notre société et affaiblit l’autorité de l’État. Ce texte est non pas une option, mais une nécessité. Mes chers collègues, adoptons le avec la conviction qu’il est encore possible de redresser notre pays, de restaurer l’autorité de l’État et de protéger ceux qui, chaque jour, défendent la République face à l’irresponsabilité de l’État. La parole

Grand. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, l’heureuse initiative de notre collègue Stéphane Demilly s’inscrit dans un contexte fort délicat. Je salue, monsieur le ministre d’État, les propos rassurants qui ont été les vôtres et qui ne seront pas étrangers à des votes qui, jusque là, n’étaient pas certains. Au cours de l’année 2023, la presse s’est fait l’écho du refus des maires Robert Ménard, de Béziers, et Stéphane Wilmotte, d’Hautmont, de procéder au mariage d’une Française avec un ressortissant algérien en situation irrégulière, de surcroît placé sous OQTF.

En l’état actuel du droit, la liberté du mariage et la régularité du séjour sont deux notions dissociées. La première n’est pas conditionnée à la seconde. La liberté du mariage peut être restreinte seulement par l’absence de consentement, la polygamie, la consanguinité et la minorité. La liberté matrimoniale constitue une liberté fondamentale à valeur constitutionnelle garantie au niveau européen par la CEDH, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Nous n’entendons pas remettre en cause ces principes. Cette proposition de loi à remédier à l’impossibilité, pour le maire, de s’opposer à un mariage dont l’un des futurs époux est en situation irrégulière et parfois, de surcroît, sous obligation de quitter le territoire national, voire, comme dans le cas de Béziers, condamné pour vol avec violence, ce qui aurait dû accélérer la mise en œuvre de l’OQTF, évitant ainsi à un maire de se retrouver devant la justice. L’article unique de ce texte crée un nouvel article

pour leurs administrés. La commission des lois a parfaitement cerné les difficultés constitutionnelles soulevées par ce texte et a tenté de les résoudre. L’idéal serait que le maire puisse saisir le préfet et le parquet dès lors que l’irrégularité du séjour est constatée, afin que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire soit accélérée ou annulée si elle n’a plus lieu d’être.

Refuser ce constat en ne luttant pas contre l’immigration illégale, c’est encourager ceux qui sont les marchands d’esclaves de notre siècle. C’est pourquoi la France doit s’attaquer à la racine du problème, et je veux saluer l’engagement du ministre de l’intérieur, Bruno Retailleau, sur cette question.

Personne en France n’est obligé de se marier pour s’aimer, sinon cela se saurait ! Les enjeux financiers de ces mariages frauduleux sont tels que certains individus n’hésitent pas à menacer l’officier d’état civil qui aurait le malheur de s’opposer à leur union. En effet, selon certains médias, les tarifs varient selon le pays d’origine : 8 000 euros quand on vient d’Afrique subsaharienne, 15 000 euros pour un Algérien ou un Tunisien et près de 30 000 euros pour un Chinois. Cela a été relaté dans la presse sans être contesté, et il y a même eu des procès. L’argent est ensuite réparti entre la filière et l’époux français. D’ailleurs, en 2021, un réseau de mariages blancs avait été démantelé

Au total, près d’une centaine d’unions frauduleuses ont été recensées en une décennie, et ce n’est là que la partie émergée de l’iceberg. De nombreux maires ont dénoncé ces pratiques, que ce soit grâce aux informations dont ils disposaient ou lors du dépôt d’un dossier de mariage pour lequel l’intention matrimoniale était jugée douteuse. aujourd’hui, certains officiers d’état civil, parce qu’ils sont trop souvent exposés et pas assez soutenus par l’État, n’osent même plus dénoncer ces mariages. Quand je suis devenue maire des XI et XII arrondissements de Marseille, j’ai alerté les autorités sur ces mariages qui, sous couvert d’un « droit à l’amour

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, il nous est demandé aujourd’hui de statuer sur une proposition de loi visant à interdire le mariage en France lorsque l’un des futurs époux réside de manière irrégulière sur le territoire français.

En outre, le droit au mariage est une liberté individuelle largement consacrée par le Conseil constitutionnel, qui a considéré, dans sa décision du 20 novembre 2003, que la liberté matrimoniale constituait une liberté fondamentale à valeur constitutionnelle. Nos collègues qui défendent cette proposition de loi ont un objectif clairement défini : faire en sorte que les maires ne soient plus tenus de célébrer l’union lorsque l’un des futurs époux ne dispose d’aucun titre de séjour valide

constitutionnelles qui s’imposent à nous. C’est la raison pour laquelle la commission des lois n’a pas adopté ce texte. En effet, nous comprenons de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qu’il est impossible pour le législateur, en l’état du droit, de subordonner systématiquement le mariage à une condition de régularité du séjour. Sa compétence réside plutôt dans l’encadrement de l’exercice de la liberté matrimoniale par des mesures visant à lutter contre les mariages frauduleux, à l’image des mariages de complaisance. Ces mariages sont conclus dans l’unique but, pour un ressortissant étranger en situation irrégulière, d’obtenir un titre de séjour. Il n’est pas acceptable qu’un individu en situation irrégulière puisse, par le biais du mariage, régulariser sa situation en France. Il n’est pas acceptable que l’institution du mariage puisse être détournée de manière frauduleuse à des fins purement administratives. Bien entendu, l’ancienne maire que je suis a déjà été confrontée à ces époux qui ne s’aimaient que sur le papier, ces époux qui ne parvenaient même pas à se témoigner le moindre signe d’affection, alors qu’ils s’apprêtaient à s’unir pour la vie… Que pouvais je faire face à ces signes évidemment suspects ? Le maire dispose bien du pouvoir légal de signalement ou d’appréciation de la validité d’une demande en mariage, mais s’opposer à un mariage l’expose à lourdes sanctions. Il n’est donc plus acceptable que les maires soient en première ligne et que leur responsabilité soit ainsi exposée. Il n’appartient pas non plus à l’officier d’état civil de juger ou de contrôler la régularité du séjour, puis de se prononcer sur la validité ou non du mariage, dans la mesure où ce n’est ni son rôle ni sa vocation. Comme je l’ai indiqué précédemment, le défaut de l’autorisation de séjour de l’un des futurs époux ne constitue pas, à lui seul, un motif suffisant d’opposition de la part du maire. En droit positif, la seule solution pour l’officier d’état civil est de suspendre un mariage présumé suspect et de saisir le procureur de la République, qui peut s’y opposer. Une évolution législative portant sur ce point précis pourrait constituer une voie de passage pertinente, afin de mieux protéger les maires. Nous soutiendrons les propositions du rapporteur qui iront en ce sens. Pour le groupe RDPI, ce texte doit donc en premier lieu protéger les maires. Alors que la France est confrontée à une importante crise de vocations chez les élus, nous devons les protéger dans ce type de situations. Nous devons leur offrir un cadre précis pour mener leur action, ainsi que des outils nouveaux, pour qu’ils puissent remplir leur rôle avec efficacité et sérénité. il est crucial de trouver un équilibre. Nous ne souhaitons pas contraindre par une interdiction absolue tous les couples dont l’un des futurs époux se trouve en situation irrégulière, surtout surtout lorsque l’absence de titre de séjour n’est que temporaire et liée à des difficultés administratives. Sur ce fondement, le droit à la vie privée et à l’établissement d’une famille ne doit pas être mis en cause. En commission, le rapporteur s’est engagé à modifier cette disposition, afin de dégager une voie de passage conforme à l’esprit du texte et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Nous soutiendrons ces amendements. La parole

d’une part, des mariages arrangés ou simulés, c’est à dire ceux dans lesquels l’un des futurs époux ou les deux ne fait pas la preuve d’une véritable intention matrimoniale ; il s’agit, d’autre part, du rôle du maire dans la procédure de refus d’un mariage.

C’est un objectif louable, qui doit, comme tous nos objectifs, être adapté au respect des droits et des libertés, ainsi qu’aux réalités pratiques vécues sur le terrain. la seconde problématique, les élus du groupe RDSE souhaitent évidemment que les maires soient protégés par la loi dans l’exercice de leur mission d’officier d’état civil. À ce titre, il me semble, eu égard à mon expérience, que les maires sont souvent bien seuls face à des situations dans lesquelles ils n’ont pas les moyens d’agir directement. Si nous souscrivons aux objectifs de ce texte, nous souhaitons affirmer notre opposition au dispositif proposé ainsi qu’à la méthode suivie. En effet, nous sommes tout à fait étonnés de nous retrouver en séance publique à discuter d’un texte dont l’inconstitutionnalité ne fait aucun doute, puisqu’il porte atteinte à la liberté du mariage. Le respect de cette liberté est protégé par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que par l’article 12 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme

s’opposent à ce que le caractère irrégulier du séjour d’un étranger fasse obstacle, par lui même, au mariage de l’intéressé ». Mes chers collègues, vous connaissez la culture de la délibération du groupe RDSE, qui promeut le dialogue, plutôt que l’opposition sans débat. Mais la délibération nécessite des règles claires, dans le respect desquelles nous pouvons aborder sereinement les sujets et,, aboutir à des décisions collégiales. En l’espèce, la discussion d’une sorte de lit de justice constitutionnel par la loi à la défaveur des libertés fondamentales fait obstacle aux conditions d’un dialogue serein. Malgré les amendements déposés qui, dans la stratégie voulue par la majorité, devraient supplanter les dispositions initiales, nous maintiendrons notre scepticisme sur la méthode. mon plein et entier soutien aux maires qui font ou ont fait face à des situations très compliquées relatives à ce sujet. Le Sénat se tient aux côtés des élus locaux pour les conforter dans leur mission au quotidien et pour modifier le cadre législatif si cela se révèle

et quelles que soient les positions des uns et des autres sur l’immigration, personne ne peut comprendre que quelqu’un qui est en situation irrégulière et qui est soumis à une OQTF puisse aller tranquillement se marier devant un maire, lui même démuni… Les maires ne sont pas démunis ! … et contraint de faire

Nous ne sommes pas l’annexe du Conseil d’État ou du Conseil constitutionnel. C’est à nous qu’il revient de faire la loi

concessions. Bravo ! La discussion générale est close. Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le groupe CRCE K a déposé cette motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité sur cette proposition de loi visant à interdire un mariage en France lorsque l’un des futurs époux réside de façon irrégulière sur le territoire. En effet, ce texte est inconstitutionnel. Je ne vous apprends rien, vous le savez et vous l’avez reconnu. Vous l’avez d’ailleurs acté lors de la réunion de la commission des lois. À plusieurs reprises, notamment dans sa décision du 20 novembre 2003, le Conseil constitutionnel a rappelé que la liberté du mariage était protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. À ce titre, le caractère irrégulier du séjour de l’un des futurs époux ne peut pas « faire obstacle en lui même » au mariage. Tel est le socle posé par la jurisprudence constitutionnelle. En plus de ce socle constitutionnel, la liberté du mariage est également garantie par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen. De plus, les sages de la rue de Montpensier rappellent que, comme toute liberté, la liberté du mariage n’est pas absolue, absolue, le législateur pouvant fixer les conditions du mariage, dans le respect des exigences de caractère constitutionnel. Notre code civil prévoit ainsi quatre limitations. Il est interdit aux personnes mineures de se marier, sauf cas exceptionnels. Les mariages polygames ou consanguins sont également interdits. Enfin, un consentement libre et éclairé est une condition indispensable à la célébration du mariage. On comprend bien l’intérêt de ces bornes. Elles se justifient par la gravité et par la dangerosité de tels comportements sur notre société et sur les individus que nous devons protéger.

de consulter le code civil : si, lors de la célébration, l’officier d’état civil a des doutes sérieux quant à la légalité d’un mariage, il saisit sans délai le procureur de la République. Ce dernier, sur le fondement d’une enquête, tranchera alors le sort de ce mariage, par décision motivée. Il y aurait ainsi, quelques centaines de cas d’opposition au mariage formulés par le procureur de la République au motif d’une suspicion de mariage simulé ou arrangé.

En donnant au procureur de la République la responsabilité de la décision quant au doute sur la légalité d’un mariage, nous protégeons le maire, officier d’état civil. En cette période de violences croissantes contre les élus, il n’est pas inutile

il encourra une peine pouvant atteindre cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, ainsi qu’une peine complémentaire d’inéligibilité. Nous ne sommes pas du côté des maires médiatiques dont l’agenda d’extrême droite est bien loin des intérêts de la France et des gens qui la composent. Nous sommes du côté de ceux qui, chaque jour, défendent la démocratie locale et les valeurs de la République. Si la situation est ubuesque pour l’extrême droite, elle n’a rien d’insensé pour ceux qui défendent la République française. Et les maires le savent,

Croyez vous réellement que vous protégerez la France en piétinant ainsi l’universalité d’un droit fondamental ? En vérité, cette proposition de loi est un leurre un écran de fumée visant à faire oublier l’absence de réponse sur des sujets autrement cruciaux sur lesquels nous sommes attendus, qu’il s’agisse de l’emploi, du logement, de la santé ou de l’éducation.

Cette instrumentalisation politicienne de l’immigration vous disqualifie, car elle révèle une forme de soumission aux logiques électoralistes les plus cyniques. À qui donnez vous donc des gages ? Notre assemblée vaut mieux que cela. La loi, qui est l’expression de la volonté générale, ne doit pas devenir le jouet de calculs partisans au mépris de l’État de droit.

lorsqu’il s’applique aux étrangers. Par exemple, s’il est interdit d’embaucher une personne étrangère sans autorisation de travail, le salarié étranger pourra solliciter un titre de séjour sur le fondement de son travail. Il lui sera demandé de fournir en préfecture des bulletins de salaire pourtant illicites. Ce salarié illégal sera tout de même protégé par le code du travail, et c’est heureux Parce que les personnes étrangères sans papiers sont des êtres humains, leur précarité administrative ne peut pas justifier une vie sans droits. La dignité humaine est pour tous ou pour personne.

à propos d’un sujet aussi essentiel, de pouvoir mener le débat à son terme dans cet hémicycle, de pouvoir discuter et échanger calmement, sereinement, sans que des contre vérités examiner et voter les amendements. Je l’ai dit tout à l’heure, j’ai déposé un texte qui se veut clair, laconique et univoque, mais qui, à l’évidence, met un vrai sujet sur la table.

reviendrait à balayer d’un revers de la main les attentes des élus municipaux. Or ce n’est pas parce que la question est difficile qu’il faut éviter le débat. En second lieu, et pour en revenir au fond de cette motion, la jurisprudence du Conseil constitutionnel, tout comme nos engagements internationaux, n’empêche pas le législateur de proposer des adaptations à la loi, notamment lorsque le contexte, comme je l’ai déjà souligné, a sensiblement évolué. La décision du Conseil constitutionnel que vous mentionnez, ma chère collègue, date du 20 novembre 2003, année durant laquelle environ 20 000 OQTF ont été prononcées. décidées pour l’année 2023. Plus de vingt ans après, la situation a profondément changé, le ministre l’a rappelé tout à l’heure. Nous nous devons, en tant que législateurs, de prendre en compte ces évolutions. Le Conseil constitutionnel suit les mêmes principes. Dans certaines circonstances, il peut préciser ou ajuster la portée des normes constitutionnelles en fonction des réalités actuelles. Cela peut se traduire par des décisions qui étendent ou restreignent certaines libertés ou certains droits fondamentaux au regard des transformations de la société. Par exemple, des décisions relevant d’une jurisprudence antérieure peuvent évoluer à la lumière d’éléments nouveaux. C’est ainsi que fonctionne notre droit, je ne vous apprends rien. Le pouvoir d’interprétation du Conseil constitutionnel garantit que la Constitution reste un instrument vivant, capable de s’adapter aux évolutions de la société. Je l’ai dit en préambule : oui, en 2003, le Conseil constitutionnel s’était fondé sur les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui protègent la liberté personnelle.

Sans ces bornes nécessaires, l’exercice de certaines libertés pourrait empiéter sur d’autres droits fondamentaux. À titre d’exemple, le principe d’égalité devant la loi est bien protégé par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le mot « Égalité » est inscrit sur le fronton des mairies. Dès lors, comment expliquer que, dans une mairie, des enquêtes sont diligentées, parce que la sensibilité personnelle de l’officier d’état civil ou les moyens municipaux y concourent, alors que dans une autre mairie, rien n’est fait ?

Monsieur Gay, quand vous déclarez que nous courons après l’extrême droite,… Oui ! … permettez moi de vous dire qu’à force de mettre des œillères dogmatiques face à de vrais problèmes, c’est vous qui faites le lit de l’extrême droite ! C’est vous qui balisez le chemin

que cela comporte en termes d’éloignement, et ne pas prendre ce risque, c’est à dire renoncer à se marier, renoncer à une liberté garantie par la Constitution. En conséquence, quelle que soit la rédaction retenue, dès lors qu’un dispositif établit une connexion entre régularité du séjour et mariage, il porte nécessairement atteinte à une liberté fondamentale.

Les maires et les officiers d’état civil seront incités à sortir de leur seule mission, la célébration des mariages, pour devenir les acteurs du contrôle de l’immigration. Or, je le redis, tel n’est pas le rôle des maires ni celui de leurs adjoints. Notre rôle, lorsque nous sommes en responsabilité, est de vérifier que le mariage est fondé sur le consentement libre et éclairé des futurs époux et le souhait d’une vie commune, conformément aux principes du mariage

moment. La parole est à Mme Valérie Boyer, pour explication de vote.

comme un stratagème pour contourner nos lois. Le garde des sceaux l’a dit et redit : le mariage doit être un droit et non un passe droit

vérité, vous avez un problème avec le fait que la Constitution, les engagements internationaux de la France et la jurisprudence du Conseil constitutionnel vous empêchent de mettre en œuvre votre projet politique

pendant lequel le procureur de la République peut surseoir à un mariage soupçonné d’être frauduleux et instaurer le principe selon lequel le silence vaut sursis au mariage. Je précise que cet amendement est compatible avec l’article unique de cette

pour avoir refusé de se rendre complices d’une fraude manifeste. Cette situation ubuesque est très justement décrite dans l’exposé des motifs de la proposition de loi de notre collègue Stéphane Demilly et dans le rapport de la commission des lois, tous deux excellents. Elle est révélatrice des injonctions contradictoires auxquelles les maires sont confrontés face à un État schizophrène. En tant qu’officiers d’état civil, les maires ont l’obligation de vérifier scrupuleusement les documents présentés par les futurs époux. En cas de doute, les dispositions de l’article L. 2122 32 du code général des d’un titre de séjour valide ou l’obligation de quitter le territoire français ne suffisent pas à empêcher la tenue d’une union. C’est une aberration ! Le rôle du Sénat est de protéger, de respecter et de soutenir le travail des maires et des agents municipaux qui signalent des contournements manifestes de la loi. la loi. Par ailleurs, le mariage n’est pas un instrument de régularisation administrative. Il s’agit non pas de stigmatiser qui que ce soit, mais de s’assurer de la sincérité de la réalité de la volonté matrimoniale des futurs époux. Je soutiens donc évidemment cette proposition de loi, ainsi que les amendements de nos collègues visant à trouver une voie de passage législative pour redonner aux maires les moyens de faire respecter la loi avec discernement et responsabilité. La parole

Ce texte est donc inconstitutionnel, comme en témoigne par ailleurs la jurisprudence du Conseil constitutionnel – rien que ça ! En proposant d’interdire à un Français de se marier avec un étranger sans papiers – et inversement –, la majorité sénatoriale s’enfonce encore un peu plus dans une forme de démagogie anti immigration.

la disposition introduite est mauvaise, car elle place le maire dans une position où il devra juger de la légalité d’un mariage. Elle fait de ce dernier ni plus ni moins qu’un acteur du contrôle de l’immigration.

en s’attaquant aux principes fondamentaux qui ont fait la grandeur de sa démocratie. La Constitution, avec laquelle vous semblez avoir tant de problèmes,

que faire du séjour irrégulier un obstacle à cette liberté est contraire à notre Constitution. Or qu’y a t il de plus français que la Constitution de la France, monsieur Hochart Nous proposons donc de supprimer cet article unique, car nous considérons que, derrière cette proposition de loi, il n’y a pas la lutte contre les mariages blancs, comme cela a été très bien expliqué, ni la lutte pour la France : il y a seulement la lutte contre ce qui a fait de la France une grande démocratie, à savoir le respect des droits fondamentaux, des libertés fondamentales et de nos engagements internationaux.

à nous, législateurs, que ce prétendu bon sens aurait désormais une valeur supérieure à la Constitution, à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à la convention européenne des droits de l’homme…

ses fonctions d’officier de police judiciaire sous le contrôle du procureur de la République. C’est donc bien ce dernier, et lui seul, qui a autorité pour faire opposition à un mariage.

Merci